Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l’inscription à l’ordre du jour du mercredi 27 novembre d’une déclaration en application de l’article 50 1 de la Constitution portant sur les négociations en cours relatives à l’accord d’association entre l’Union européenne et le Mercosur, suivie d’un débat et d’un vote. Ce débat pourrait avoir lieu à seize heures trente, à l’issue des questions d’actualité au Gouvernement. Acte est donné de cette demande. Pour ce qui concerne son organisation, nous pourrions prévoir que les orateurs des groupes interviennent selon un ordre suivant l’effectif décroissant des groupes, avec les temps de parole suivants : quatorze minutes pour le groupe Les Républicains, douze minutes pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, dix minutes pour le groupe Union Centriste, minutes pour les autres groupes, trois minutes pour un sénateur non inscrit. Le délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat serait fixé au mardi 26 novembre, à Y a t il des observations ?… Il en est ainsi décidé. Nous reprenons la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’amendement n° 575 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l’article 7.

et toujours dans l’attente d’une loi Grand Âge, qui nous permettrait d’avoir une vision générale des exonérations en fonction des différents statuts des établissements, ainsi que de répondre aux professionnels toujours oubliés du Ségur, je vous propose cet amendement qui vise à assurer le financement de la branche autonomie en assujettissant à la contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) des revenus qui en sont aujourd’hui exonérés, notamment les sommes allouées aux salariés au titre de l’intéressement, de la participation de l’employeur au plan d’épargne, ainsi que les revenus des travailleurs indépendants. Il s’agit donc d’élargir l’assiette de la CSA, qui est actuellement limitée aux cotisations patronales d’assurance maladie.

à la charge unique des employeurs. Il ne semble donc pas souhaitable d’alourdir les cotisations des travailleurs indépendants, qui bénéficient en contrepartie d’une moins bonne couverture, vous en conviendrez, mes

Cet amendement vise à créer une contribution de 1 % assise sur les revenus des capitaux mobiliers, pour financer la cinquième branche de la sécurité sociale, ainsi que le préconise le rapport Vachey. La création de la branche autonomie n’a pas donné lieu à un financement pérenne de la perte d’autonomie ; or le rapport or le rapport Libault fait état d’un besoin de financement annuel de 6 milliards d’euros à partir de 2024 et de 9 milliards d’euros à partir de 2030. Il apparaît donc nécessaire de doter cette cinquième branche de financements propres pour permettre son équilibre et une montée en charge progressive de sa capacité financière. la création d’une contribution sur les dividendes versés aux actionnaires constituerait un risque réel pour l’attractivité de la place financière française

Monsieur le ministre,

Briante Guillemont. Depuis la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie, la CNSA a été chargée de répondre aux défis du vieillissement de la population. Cependant, cette cinquième branche nécessite des financements pérennes et ambitieux. Dans un contexte d’inégalités patrimoniales croissantes, il semble juste que les efforts financiers pour soutenir l’autonomie soient partagés, en mobilisant une partie des transmissions de patrimoine les plus importantes. Aussi, cet amendement vise à créer une contribution sur les transmissions de patrimoine qui ne s’appliquerait qu’aux successions et donations dont l’actif net taxable dépasse 150 000 euros par bénéficiaire. Le taux de cette contribution a été fixé à 1 % sur l’excédent au delà de ce seuil. L’intégralité des fonds générés par cette mesure sera directement allouée à la CNSA.

entraîne un prélèvement. Le gain de la taxation existante est donc très limité par rapport à l’assiette globale, comme l’a souligné en 2021 la direction générale du Trésor : les droits de succession n’ont rapporté que 12,6 milliards d’euros L’idée d’une taxation des successions n’est pas nouvelle. Une note du Conseil d’analyse économique (CAE) de 2021 proposait déjà une réforme en profondeur de la taxation de l’héritage, laquelle permettrait de réduire les droits de succession pour 99 % de la population,

pour un rendement de 500 millions d’euros au bénéfice de la branche autonomie. Ce financement pourrait ainsi, en plus de constituer une mesurette de redistribution du patrimoine, financer en partie les besoins de cette branche, que le rapport Libault, je le rappelle, a chiffrés à 6 milliards d’euros

De plus, une telle contribution sur la transmission de patrimoine ne semble pas souhaitable : elle remettrait en cause les efforts réalisés depuis plusieurs années afin de favoriser la solidarité intergénérationnelle au bénéfice des plus jeunes.

au financement de la branche autonomie, en particulier à celui de la prise en charge à 100 % des fauteuils des personnes en situation de handicap. Vous l’aurez compris, il s’agit là d’un projet alternatif

qui repose sur les salariés, les retraités et les malades. Pourquoi les actionnaires ne participeraient ils pas, de manière symbolique, au financement de la branche autonomie pour laquelle, je le rappelle, il n’existe pas de contribution des employeurs ? Quel

La sécurité sociale a un réel besoin de financement. Cet amendement vise à dégager de nouvelles recettes en mettant à contribution les revenus financiers des entreprises.

en l’état des comptes de la sécurité sociale, la mise à contribution du capital n’est pas plus incongrue que la fiscalisation de la TVA. La CSG sur les revenus de placement est même assez proche de la philosophie de cette proposition. La seconde partie du dispositif de cet amendement est la plus importante : elle tend à moduler le taux de cotisation en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses. modulation des cotisations sociales patronales nous apparaît comme un vecteur pour encourager le développement d’une gestion vertueuse d’entreprises émancipées de la finance et porteuses d’emplois. évoluer les cotisations patronales en fonction des politiques d’emploi et de salaire menées par les entreprises au sein d’une même branche d’activité, il devient possible de peser sur leurs choix de gestion.

Au delà du cas d’Orpea mis en lumière par de Victor Castanet, nous constatons une montée en puissance des groupes privés dans le secteur des Ehpad. Entre 1986 et 2015, le nombre de places en établissements médico sociaux médicalisés a augmenté de 85 tandis que les places dans le secteur privé lucratif ont bondi de 560 %. Aujourd’hui, les cinq plus grands groupes français d’Ehpad privés sont contrôlés par des fonds de capital investissement. Cette financiarisation, encouragée par la quête de profit des investisseurs, s’est installée sous les yeux des pouvoirs publics, souvent pris de court. Les chiffres sont éloquents : les fondateurs d’Orpea détiennent aujourd’hui un patrimoine de plus de 1 milliard d’euros et les grands groupes d’Ehpad figurent parmi les 500 plus grandes fortunes françaises.

annuel représente environ 40 % du chiffre d’affaires des Ehpad privés à but lucratif. Face à cette situation, il est impératif de mieux redistribuer ces superprofits en prévoyant une contribution additionnelle affectée à la CNSA, qui permettrait de réinjecter ces excédents dans l’amélioration des soins, le soutien au personnel et une prise en charge plus digne de nos aînés. Il s’agit d’un enjeu de justice sociale et de responsabilité collective.

également tous d’accord sur la nécessité de trouver des financements pour l’autonomie, pour l’accompagnement des personnes âgées ou handicapées et pour la petite enfance.

Cette hausse viendra augmenter les ressources de la CNSA. Les départements se félicitent sur le principe de l’octroi de ces moyens supplémentaires, à l’heure où ils sont durement confrontés à un effet ciseaux entre les évolutions respectives de leurs ressources et de leurs dépenses. En conséquence, une partie de cette somme devrait leur bénéficier afin de poursuivre les politiques conduites auprès des personnes âgées. En 2024, alors que la CNSA a bénéficié d’un transfert de 0,15 point de CSG, et à l’exception d’un complément de 150 millions d’euros prévu dans le cadre de

respectivement 40 % et 30 % en moyenne – est désormais insuffisant pour faire face aux enjeux des politiques de soutien à l’autonomie, liés notamment au virage domiciliaire et au choc démographique. Il convient de rehausser en urgence ces concours pour les porter à 50 %, ce qui impliquerait une hausse des ressources de 1,4 milliard d’euros environ.

l’espérance de vie augmente et il faut que les Français puissent travailler un peu plus, d’autant qu’ils entrent plus tard dans la vie active. De plus, nous sommes confrontés aussi à la concurrence internationale, de sorte que nous avons besoin d’entreprises qui soient particulièrement performantes.

50 000 emplois. Il est impératif de disposer de 2,5 milliards d’euros supplémentaires par an. L’instauration d’une seconde journée de solidarité permettrait ce financement et montrerait une cohésion

C’est le sens de l’Histoire que d’augmenter le temps du travail pour que notre pays soit mieux armé pour affronter la compétition économique dans le monde. Allons y, n’ayons pas peur

payée par les entreprises, afin de ne pas laisser les salariés et les retraités financer, seuls, la branche autonomie. Il s’agit donc de faire participer les entreprises au financement de cette

et à la casse des droits collectifs proposée par la majorité sénatoriale. Il est possible d’augmenter la contribution des entreprises pour financer la branche autonomie sans imposer aux travailleurs de travailler gratuitement, sept heures de plus par an, comme le propose la majorité gouvernementale du Sénat. L’amendement

souscrivons à l’objectif de renforcer les moyens alloués à l’autonomie de manière pérenne, mais la quotité proposée risquerait de compromettre le consentement des travailleurs.

Par ailleurs, la proposition de la commission vise à financer la branche autonomie de la sécurité sociale pour sécuriser son avenir, en affectant une partie des recettes nouvelles directement aux départements. Nous risquerions de brouiller le message si nous allions plus loin.

Une garantie sur le taux de couverture des dépenses départementales au titre de l’APA et au titre de la PCH est notamment prévue. Nous pourrons alors débattre plus précisément de ce sujet et du financement de ces différentes prestations assurées par les départements.

au moins de manière transitoire. Deux minutes par jour,

les femmes gagnent 24 % de moins que les hommes, à compétences égales, et ce malgré les obligations instaurées par les lois Auroux de 1982. Les entreprises sont dans l’illégalité depuis quarante ans sans que cela choque personne, ou presque.

Elles représentent 99 % des assistants maternels et 97 % des aides à domicile. Elles aiment leur métier, mais elles ne parviennent pas à en vivre.

Le travail à temps partiel est donc profondément sexiste ; nous devons infléchir les pratiques des entreprises qui abusent des contrats précaires. Nous proposons d’œuvrer en faveur de l’égalité salariale et de réduire le temps partiel subi en majorant de 10 % les cotisations employeur des entreprises de plus de vingt salariés comptant dans leurs effectifs au moins 20 % de salariés à temps partiel. l’avis de la commission ?

de s’attaquer à ceux que l’on ne connaît pas ! D’une part, l’article revient sur l’exonération de CSG et de CRDS dont bénéficient les Français établis dans l’espace économique européen et en Suisse. Sur le plan juridique, cette disposition est purement et simplement inapplicable. En effet, cette exonération a été instaurée en 2015 à la suite de la condamnation de la France par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui a jugé le prélèvement de ces deux contributions incompatible incompatible tant avec l’interdiction du cumul des législations applicables en matière de sécurité sociale qu’avec la libre circulation des travailleurs. Mes chers collègues, vous conviendrez que la législation française est tenue d’être en conformité avec le droit européen. Dès lors, comment voter cet article ? Sur le plan politique, je m’y oppose fermement : j’ai même défendu, hier, un amendement qui en était l’exact contraire. Il n’aurait été que pure justice que l’ensemble des Français de l’étranger soient exemptés D’autre part, cet article prévoit que les certificats de vie nécessaires à la perception des pensions de retraite soient délivrés uniquement par les consulats. C’est méconnaître la réalité que nous vivons à l’étranger.

Dans certains pays, ces déplacements sont coûteux, parfois dangereux, voire impossibles. Pour toutes ces raisons de bon sens, le groupe socialiste propose la suppression de cet article. Je suis saisi

d’un tel dispositif favoriserait une politique du soupçon envers les étrangers, dont la contribution sur le sol français est oubliée au profit d’une focalisation sur la figure du fraudeur.

Par ailleurs, une expérimentation de la Cnav est déjà en cours dans certains pays, comme l’Algérie et le Maroc. Ainsi le dispositif proposé doublonnerait il une initiative existante en alourdissant inutilement le travail consulaire. Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer l’article

n° 1175 rectifié. Monsieur le ministre, il est vraiment regrettable, comme l’ont dit mes collègues, que l’Assemblée nationale ait adopté des dispositions présentant les retraités français comme étant des nantis et des fraudeurs. Notre amendement vise purement et simplement à supprimer l’article 7, qui assujettit les retraités à la CSG et impose l’authentification des certificats de vie par les consulats.

La seconde limite la possibilité, pour ces retraités, de s’acquitter de l’obligation qui leur incombe de justifier annuellement de leur existence auprès du GIP Union Retraite afin de pouvoir continuer à percevoir leur pension.

depuis juin 2024, par l’utilisation de données biométriques : les retraités reçoivent, de la part du GIP Union Retraite, un QR code qui leur permet de télécharger une application sur leur smartphone et d’y verser des vidéos et des photos d’eux, ainsi que des données de leurs pièces d’identité biométriques. L’Assemblée nationale a souhaité préciser dans la loi que les certificats de vie doivent nécessairement être délivrés par le consulat français. Cette précision doit permettre de lutter contre la délivrance de faux documents par des notaires ou des officiers corrompus.

Cela est contraire au droit européen, qui interdit que des personnes résidant dans un État membre et affiliées à un système de protection sociale ne cotisent à perte auprès d’un autre système de protection sociale d’un autre État membre.

ni compris. Je voudrais donc vous rappeler pourquoi il est aujourd’hui crucial d’apporter un soutien pérenne à la CFE et de sortir de l’immobilisme. Cette caisse assure une véritable mission de service public en offrant une couverture sociale à tous les Français vivant à l’étranger, sans discrimination liée à l’âge ou ou à l’état de santé. Elle incarne une solidarité universelle envers les plus fragiles grâce à la « catégorie aidée ». Pour accomplir une telle mission sociale, la CFE compte essentiellement sur les recettes provenant de ses contrats d’adhésion, conformément à l’obligation d’autonomie financière dont elle fait l’objet. De fait, contrairement aux caisses primaires d’assurance maladie, elle ne bénéficie d’un soutien de l’État que pour la « catégorie aidée », mais non de taxes affectées ni de fractions de CSG.

un amendement identique a été rejeté par le Sénat l’année dernière. La commission ne connaît pas suffisamment la situation de la CFE, qui n’est pas un organisme obligatoire de sécurité sociale, pour savoir s’il est pertinent de majorer ainsi ses recettes. En revanche, il ne convient certainement pas de réduire les ressources du FSV dans le contexte actuel, alors que le PLFSS prévoit pour la branche vieillesse un déficit croissant jusqu’en 2028. Par ailleurs, l’amendement n° 1218 du Gouvernement, que nous examinerons un peu plus tard,

calculées selon les seuils applicables aux entreprises de moins de onze salariés. Cependant, la disposition visée prévoit également un transfert des effectifs vers les entreprises utilisatrices à partir de 2026, ce qui alourdit la gestion administrative.

d’éviter des coûts inutiles pour l’administration, et à garantir la pérennité des avantages sociaux pour les petites entreprises

Les salariés mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice par un groupement d’employeurs ne seraient comptabilisés ni dans les effectifs du groupement d’employeurs ni dans ceux de l’entreprise utilisatrice. Une telle mesure serait non seulement injustifiée,

Quant au manque à gagner total lié au travail dissimulé, il serait compris entre 8 milliards et 10 milliards d’euros, sachant que 10 % seulement des sommes redressées au titre de la lutte contre le travail dissimulé sont recouvrées, de nombreuses entreprises

dans notre pays. L’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a prévu l’obligation pour les plateformes numériques de collecter et de verser les cotisations sociales des microentrepreneurs utilisateurs des plateformes par un calcul et un prélèvement directs

visant à réformer la collecte des cotisations sociales des microentrepreneurs des plateformes numériques. L’enjeu est en effet important : la sous déclaration des revenus générés par ces activités a été soulignée, dans une note de décembre 2022, par le Haut Conseil du financement de la protection sociale,

par l’assurance maladie des informations relatives à cette fraude à l’employeur de l’assuré concerné. Ainsi, sur le fondement de cette disposition légale, en cas de délivrance de délivrance frauduleuse d’un arrêt de travail ou d’exercice d’une activité non autorisée pendant l’arrêt maladie, la caisse primaire d’assurance maladie constatant la fraude serait habilitée à porter cette information à la connaissance de l’employeur.,

pour objet de contrôler les déplacements aériens, est autorisé par la loi à titre expérimental. Il est accessible aux agents des ministères de l’intérieur, de la défense et des transports ainsi qu’à ceux des douanes, pour les besoins liés à la prévention de certaines infractions qui concernent les actes de terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation.

Le droit est clair : les personnes en situation irrégulière ne peuvent bénéficier d’aucune prestation sociale, à l’exception de l’aide médicale de l’État (AME) et de l’accès à un hébergement d’urgence.

Monsieur le ministre,

? Sont inscrites au fichier des personnes recherchées les personnes qui font l’objet de décisions judiciaires devant être exécutées, celles qui sont recherchées dans le cadre d’une enquête pénale

? Prévue à l’article L. 133 1 du code de la sécurité sociale, la procédure de flagrance sociale permet aux organismes de recouvrement, lorsque la situation et le comportement de l’entreprise ou de ses dirigeants met en péril le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues, de dresser un procès verbal sur la base duquel le directeur de l’organisme peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de saisir les biens de l’entreprise. Les fraudes aux prestations sont toutefois généralement commises non par des entreprises, mais par des particuliers. Un procès verbal n’est pas nécessaire pour constater une telle fraude, tandis que le problème principal en la matière réside non pas dans la capacité des Urssaf à saisir les biens du fraudeur, mais dans la fréquente insolvabilité de celui ci. Il ne paraît donc pas judicieux d’étendre la flagrance sociale au delà des cas de travail dissimulé. Avis défavorable.